? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai pris acte de la démission, à compter du mercredi 4 octobre 2017 à minuit, de M. Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne.

Son siège devenu vacant sera pourvu par une élection partielle. Je profite de cette occasion pour remercier devant vous Jean-Pierre Raffarin pour l'exercice de son mandat de sénateur,

J'informe le Sénat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 L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission des affaires européennes. Conformément à l'article 73 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe a été publiée. Cette liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.